La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Rendre la République forte et efficace », telle fut la volonté du général de Gaulle.

qu'il existe, au-dessus des luttes politiques, un arbitre national, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, que le Parlement et le Gouvernement collaborent mais demeurent séparés quant à leurs responsabilités. Telle est la structure équilibrée que doit revêtir le pouvoir. » En soixante années, marquées par des crises économiques, sociales et politiques, nos institutions ont toujours résisté aux chocs. Après quatre alternances politiques et trois cohabitations, notre Constitution a fait la démonstration de sa solidité. Je pense également à la fin du processus de décolonisation, à la crise de mai 1968, ou encore, si près de nous, aux terribles événements qui frappent notre pays depuis janvier 2015. l'heure où certaines des grandes démocraties européennes, d'ailleurs fondatrices de l'idée d'union, connaissent l'instabilité, notre Constitution est une chance pour notre pays. En 1958, en pleine crise institutionnelle, il fallait remédier à l'instabilité gouvernementale de la IV République qui paralysait le pays alors qu'il était confronté à des défis majeurs. La nouvelle Constitution allait donc renforcer le pouvoir exécutif et rompre avec ce que l'on qualifiait de « régime des partis » pour rendre l'action publique plus efficace. Le Président de la République est devenu un arbitre, tel que défini par le discours de Bayeux, au-dessus des partis politiques, et il dispose de compétences propres. Après la révision constitutionnelle de 1962, il a eu la légitimité du suffrage universel direct. À vingt-quatre reprises, notre Constitution a été révisée, pour renforcer l'État de droit et les pouvoirs du Parlement avec l'élargissement, en 1974, des modalités de saisine du Conseil constitutionnel, pour se conformer à nos engagements européens et internationaux- je pense notamment au traité de Maastricht, en 1992 -, pour consacrer le caractère décentralisé de notre République et les libertés locales, en 2003, ou encore pour marquer notre attachement à certaines valeurs- je pense à la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort, en 2007. Au fil du temps temps et de la pratique, mais aussi avec le passage au quinquennat et avec l'inversion du calendrier électoral, les équilibres de la V République ont évolué. Pour reprendre la citation du sage Solon, à laquelle le général de Gaulle faisait référence à Bayeux, « quelle est la meilleure Constitution ? Dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. Il s'est donc avéré nécessaire d'adapter notre système institutionnel pour rééquilibrer les pouvoirs. La meilleure illustration de cette adaptation est la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V République, issue des travaux de la commission dite Balladur : un pouvoir exécutif mieux contrôlé, un Parlement renforcé et des droits nouveaux pour les citoyens. Mes chers collègues, renforcer les prérogatives du Parlement est en réalité indispensable à notre démocratie. Un gouvernement qui ne rend pas de comptes aux représentants du peuple, un gouvernement qui n'est pas régulé dans sa production législative est un gouvernement contestable. Montesquieu l'exprimait Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Préserver les pouvoirs du Parlement, c'est préserver les fondements de la démocratie représentative. Affaiblir le bicamérisme, c'est affaiblir tout le Parlement. L'un des fondements de la V République, c'est, quoi que l'on ait dit et malgré les vicissitudes de l'histoire, le bicamérisme au coeur du discours de Bayeux : « Il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets revient à une assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entières. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. Le dialogue bicaméral et la navette parlementaire, à laquelle je suis tellement attaché, comme je suis attaché à la commission mixte paritaire, sont des conditions de la qualité de la loi. Nous devons nous employer Nous devons nous employer à ce que le Sénat, représentant les collectivités territoriales de la République, continue à incarner, par sa composition, l'ensemble des territoires de notre pays. Sous prétexte de réduire le nombre de parlementaires, on ne doit pas condamner au quasi-silence certains territoires de notre pays dont la démographie serait plus faible. Ce lien avec les Ce lien avec les territoires confère aussi au Sénat un autre atout : la proximité avec les élus locaux, tous les élus locaux, qui, à l'heure de la mondialisation, constituent l'un des socles fondamentaux de la cohésion nationale. Il n'est pas de République forte sans institutions puissantes » : je partage ce constat fait par le Président de la République, Emmanuel Macron, devant le Congrès, en juillet 2017. La révision constitutionnelle devra donc s'inscrire dans la continuité de celle de 2008. Elle doit avoir pour objectif de mieux faire la loi, de réconcilier nos compatriotes avec leurs parlementaires et de préserver la représentation des territoires. Le pouvoir constituant appartient au Parlement. Le Sénat a des propositions solides à faire ; je crois qu'il sera au rendez-vous. Réformer la France est difficile, mais réviser la Constitution ne l'est pas moins. Il n'est pas facile de distinguer entre l'intangible et ce qui doit être modernisé ni de résister à la pression de l'opinion publique tout en tenant compte de son aspiration au changement. Le général de Gaulle, lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964, expliquait qu'« une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. » Il me paraît primordial de se souvenir de ce triptyque pour replacer au coeur du contrat républicain le renforcement indispensable de la confiance de nos concitoyens dans la République. La place du Parlement au sein de nos institutions n'est pas un sujet mineur. Elle engage toute notre conception de l'équilibre entre les pouvoirs. Un anniversaire, c'est l'occasion de réfléchir à nos fondamentaux, à leur nécessaire évolution lorsque la société change,

en tête le drame qui s'est déroulé cet été en Italie. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat, lors de sa séance du mardi 25 septembre 2018. La commission des lois a déclaré cette demande conforme aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance

En conséquence, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission d'information.

dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur du débat disposera d'un temps de parole de huit minutes ; puis le Gouvernement

s'est traduit par un décret et par plusieurs arrêtés publiés le 16 juillet dernier. Les élèves entrés cette année au lycée constitueront la première cohorte concernée ; ils passeront les épreuves terminales dans leur nouveau format en 2020 et en 2021. Comme le soulignait notre collègue Max Brisson, auteur avec Françoise Laborde d'un excellent rapport sur le métier d'enseignant, le caractère restrictif du domaine de la loi en matière d'éducation a pour conséquence que le Parlement, au-delà du vote des crédits, est davantage amené à se pencher sur des questions de faible importance- par exemple, les modalités d'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires -plutôt que sur des questions de fond comme celle qui nous réunit cet après-midi. cet après-midi. Ainsi la commission a-t-elle souhaité la tenue de ce débat en séance publique, afin d'évoquer avec vous, monsieur le ministre, et sous le regard de nos concitoyens, les enjeux de cette réforme, et d'obtenir des réponses aux questions que mes collègues vous poseront. bien sûr mobilisés Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis des crédits de l'enseignement scolaire, et Laurent Lafon, qui a défendu les amendements de notre commission sur l'orientation scolaire à l'occasion de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Commençons par reconnaître, monsieur le ministre, que vous avez eu, avec la confiance du Gouvernement, le courage de vous attaquer à un sujet d'envergure, sur lequel nombre de vos prédécesseurs avaient échoué ou auquel monument national » et rite initiatique pour les jeunes lycéens, pose, sous sa forme actuelle, un certain nombre de questions, dont la première réside dans sa finalité, dans la mesure où, s'il ouvre les portes de l'enseignement supérieur, il n'intervient qu'après l'affectation

Nous partageons votre ambition d'un baccalauréat plus simple, mais non moins exigeant, et comportant moins d'épreuves terminales, sans toutefois renoncer à un tronc commun, garant d'une culture générale nécessaire à une citoyenneté éclairée.

La fin des séries dans la voie générale est une très bonne chose ; les combinaisons d'enseignements de spécialités donneront aux élèves une plus grande liberté de choix et leur permettront de construire des parcours de formation adaptés à leurs goûts et à leurs ambitions.

l'allégement des emplois du temps, l'accompagnement renforcé pour l'orientation dès la classe de seconde, ou encore la prise en compte, à hauteur de 40 % de la note finale, des notes obtenues tout au long de l'année, ce qui permet de récompenser la constance et la rigueur dans le travail. Si nous en soutenons les principes et les orientations, les modalités de la réforme et les conditions de sa mise en oeuvre posent néanmoins un certain nombre de questions- je n'en citerai que quelques-unes. La première porte sur les modalités du contrôle continu. Dans un souci d'équité entre les élèves et les établissements, les trois quarts de la note de contrôle continu proviendront d'épreuves dites « communes », organisées dans un cadre très contraignant qui rappelle furieusement le baccalauréat actuel. Ces épreuves, se déroulant au cours des années de première et de terminale, prendront appui sur une banque nationale de sujets, les copies étant anonymes et corrigées par d'autres professeurs que ceux de l'élève. Dans ces conditions, l'allégement annoncé de l'organisation pourra-t-il vraiment être pourra-t-il vraiment être atteint, dans la mesure où les établissements seront contraints d'organiser régulièrement des « mini-baccalauréats » qui empiéteront sur le temps d'enseignement ? Autre sujet de préoccupation pour les membres de la commission : comment s'articulera le futur baccalauréat avec Parcoursup ? Afin que le baccalauréat conserve tout son sens, il me semble important que les notes obtenues soient prises en compte, dans la plus large mesure possible, dans l'affectation dans l'enseignement supérieur. Or, vous l'avez annoncé, monsieur le ministre, les épreuves terminales auront lieu au retour des vacances de printemps, soit bien trop tard pour que les résultats soient pris en considération dans Parcoursup. Il semble que vos discussions avec le ministère de l'enseignement supérieur soient encore en cours ; êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous dire quand auront lieu les épreuves terminales ?

Si l'on peut aisément concevoir une forme de spécialisation des lycées autour de certains enseignements en ville, il en va autrement en milieu périurbain et dans le monde rural, où les élèves n'ont souvent qu'un lycée de secteur. Il serait regrettable que les élèves des territoires ruraux soient privés de la possibilité de choisir leurs enseignements du seul fait que leur lycée ne propose pas les matières désirées, d'autant qu'avec le jeu des « attendus » de Parcoursup, ils seront désavantagés pour suivre les études de leur choix. Vous savez, monsieur le ministre, combien notre assemblée est attachée à l'équité territoriale ; la ruralité ne doit pas être oubliée ni défavorisée.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est évidemment avec grand plaisir que je viens échanger avec vous sur la question du baccalauréat. d'un sujet dont a déjà discuté le Sénat à l'occasion de différents débats que nous avons eus précédemment, mais nous avions en quelque sorte rendez-vous, rendez-vous qui a lieu aujourd'hui, pour approfondir tout ce qui touche au baccalauréat.

en réformant le baccalauréat, nous voulons que, en le préparant, les élèves préparent ce qui les fera réussir après. En d'autres termes, nous voulons en finir avec une certaine artificialité de l'exercice,

au moment des admissions dans l'enseignement supérieur. La question des calendriers sera donc réglée dans un sens qui permettra une telle prise en compte des disciplines de spécialité. Le Premier ministre avait précisé, dès sa déclaration de politique générale, que la première session de ce nouveau baccalauréat interviendrait en 2021 et qu'elle concernerait donc les élèves entrés en classe de seconde Le Président de la République lui-même avait pris au cours de la campagne présidentielle des engagements sur la structuration de ce nouveau baccalauréat, notamment sur la question du contrôle continu et des épreuves anticipées. Après une consultation conduite par M. Pierre Mathiot, à qui j'avais confié cette mission, puis une concertation que j'ai menée personnellement avec les partenaires de l'éducation nationale, nous avons, au mois de février dernier, présenté une réforme

Nous renouvelons donc à la fois les contenus, les contours et les volumes horaires de cette discipline, qui est affichée comme un moment clef en fin de parcours.

pour valoriser la régularité du travail des lycéens, donc pour contribuer à en finir avec le bachotage que j'ai évoqué, il y aura une grande part de contrôle continu, qui représentera quelque 40 % de la note finale.

Ces épreuves communes auront évidemment de l'importance pour souligner la régularité du travail de l'élève.

Les élèves ne joueront donc plus leur examen sur une seule semaine d'épreuves. L'organisation sera mieux répartie sur les classes de première et de terminale. Elle ne paralysera plus les lycées en fin d'année scolaire. Aussi, le baccalauréat de 2021 sera à la fois pleinement national, pleinement juste et pleinement facteur de réussite.

aux élèves de seconde qui auraient des bases fragiles. À partir de la rentrée de 2019, l'implantation des spécialités permettra d'accompagner au mieux les élèves, de les soutenir dans leur parcours et d'organiser

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé. Dans le débat interactif, la parole est à M. Pierre Ouzoulias. Madame la présidente, madame la présidente de la commission, monsieur le ministre, malgré les réformes législatives récentes, le premier cycle de l'enseignement supérieur demeure ouvert à tous les titulaires du baccalauréat, qui en constitue toujours le premier diplôme.

qui souhaitent que les résultats du baccalauréat soient mieux valorisés dans ce dispositif nouveau. Le diplôme du baccalauréat conserve l'avantage d'être national et anonyme, c'est-à-dire de donner les mêmes droits à tous les candidats, quel que soit leur lycée d'origine et indépendamment des facilités procurées par leur milieu social. La ministre en charge de l'enseignement supérieur semble avoir entendu cette requête, puisqu'elle a récemment déclaré étudier une réforme de Parcoursup pour rendre les dossiers plus anonymes. Néanmoins, dans le même temps, Mme Vidal a annoncé, sans doute à l'issue d'une concertation interministérielle intense, que le calendrier de Parcoursup serait considérablement resserré, pour que les inscriptions administratives soient réalisées avant la fin du mois de juillet. Cela rend matériellement très difficile l'intégration de tous les résultats du baccalauréat, sauf à réduire drastiquement le temps d'examen des dossiers par les établissements de l'enseignement supérieur. Cette réforme du calendrier de Parcoursup est peu compatible avec votre volonté de maintenir le statut du baccalauréat, Au-delà de cette divergence ministérielle sur le calendrier, je veux vous interroger sur le rôle pédagogique et légal que le Gouvernement veut donner à ce diplôme pour clore le cycle des études secondaires et ouvrir celui des études supérieures. La

les premiers effets de la réforme du nouveau baccalauréat de 2021 vont se faire sentir dès cette année scolaire 2018-2019. En effet, les lycéens qui sont entrés cette année en classe de seconde devront faire un choix au troisième trimestre pour leur passage en première. La réforme du baccalauréat que vous présentez, monsieur le ministre, met en place un examen resserré autour de quatre épreuves écrites, dont le français et la philosophie, et d'un grand oral. Elle supprime les séries L- littéraire -, ES- économique et sociale -et S- scientifique -dans la voie générale. À la place, les lycéens choisiront trois matières principales, appelées « spécialités », puis deux seulement en terminale, qui feront l'objet d'épreuves écrites finales. En outre, la réforme prévoit une dizaine de spécialités, depuis « art » jusque « numérique et sciences informatiques », en passant par « langues et littératures étrangères Monsieur le ministre, tous les établissements pourront-ils proposer la totalité de l'offre et les lycéens vont-ils vraiment pouvoir choisir librement les trois matières, en panachant des disciplines scientifiques avec d'autres, plus littéraires, ou bien va-t-on avoir des triplettes toutes faites et imposées ? Je crains qu'il n'y ait un important hiatus entre le discours généreux qui a mis en avant le choix des élèves et la réalité contrainte que l'on commencera à connaître au début de l'année 2019 ... Comment informer et conseiller les jeunes dans leur orientation si l'on ne connaît pas déjà le contenu des disciplines que le Conseil supérieur des programmes doit finaliser avant le début de l'année 2019,

Enfin, comme l'a dit mon excellent collègue Pierre Ouzoulias, n'a-t-on pas fait les choses dans le désordre en lançant Parcoursup dès la rentrée de 2018, avant la réforme du bac de 2021 ? La parole

Vous verrez, si vous ne le voyez déjà, qu'il existe une très grande cohérence entre le baccalauréat qui se profile et Parcoursup, dans une vision « lycée-licence » que nous assumons bien sûr pleinement.

Les inquiétudes soulevées par les personnels de l'enseignement agricole et les premières annonces permettent d'en douter. L'agronomie devient une option facultative, alors qu'elle était un enseignement de spécialité obligatoire. Cette situation est inquiétante quand on sait que les titulaires d'un baccalauréat scientifique obtenu en lycée agricole se destinent souvent à devenir ingénieurs agronomes. Le choix de seulement deux spécialités en terminale est problématique quand la poursuite d'études supérieures en requiert trois, comme en classe préparatoire et sciences de la vie et de la terre, ou SVT. Par ailleurs, certains lycées agricoles ne seront pas en mesure de proposer tous les binômes de disciplines et, face à ce risque, les parents risquent de préférer les lycées privés. La question de la survie du service public de l'enseignement agricole est donc clairement posée. Concernant le baccalauréat sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, ou STAV, seul baccalauréat technologique de l'enseignement agricole, il sera modifié, sans que l'on dispose de La réforme laisse planer le risque d'une diminution d'horaires, donc d'un appauvrissement des contenus. Pouvez-vous nous en préciser les contours ? Par ailleurs, la filière de l'enseignement agricole, seule à être placée sous la responsabilité du ministère de l'agriculture, aurait été oubliée dans les choix proposés par Parcoursup. C'est grâce à la vigilance des enseignants que les filières proposées par les établissements agricoles ont été ajoutées. Certes, la double tutelle de cet enseignement ne simplifie pas les choses, mais comment mieux prendre en compte ces spécificités lors des réformes de l'éducation

La parole est à Mme Colette Mélot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, simplifier l'organisation d'un examen bicentenaire et mieux armer les bacheliers dans la perspective de leurs études est un objectif que nous ne pouvons que saluer, d'autant qu'il répond aux attentes de la plupart des acteurs du monde éducatif, favorables à une évolution de ce qui s'apparente aujourd'hui à un rite de passage. L'examen reste la clef d'entrée vers le supérieur, mais la situation est paradoxale : les taux de réussite du baccalauréat frôlent les 90 alors que nombre de bacheliers échouent ensuite à l'université. Sa sélectivité est désormais remplacée par le jeu des mentions et des filières. La convoitée mention « Très bien » est le nouveau sésame pour franchir la porte des établissements les plus prestigieux. Il y a non plus un bac, mais des bacs. Aussi le baccalauréat, ce « quelque chose d'incroyablement antique » décrit par Sartre, mérite-t-il cette nouvelle réforme, positive en bien des points. Monsieur le ministre, je souhaite aujourd'hui mettre l'accent sur le grand oral, qui remettra à l'honneur une capacité fondamentale, que chacun doit maîtriser au plus tôt savoir s'exprimer en public de façon claire et intelligible. Cet oral dit « de maturité » sera préparé dès la classe de première et viendra valider la capacité du lycéen à mener un projet qui lui est propre et son aptitude à le vendre face à un jury. Les compétences recherchées répondent également aux besoins du marché du travail et de l'économie. Aujourd'hui, on attend du futur salarié non seulement qu'il soit apte à s'exprimer correctement en public, mais aussi qu'il soit capable de mener à bien une réalisation personnelle. monsieur le ministre, et c'est l'objet de ma question, le futur grand oral du bac est une bonne initiative à condition d'y mettre les moyens : formation des enseignants aux techniques oratoires, heures spécifiques dédiées à leur apprentissage dans l'emploi du temps scolaire, valorisation de la parole de l'élève pendant les cours ... J'y ajoute les dispositions relatives aux élèves qui présentent un handicap. Pouvez-vous donc nous décrire les moyens que vous comptez déployer pour que ce projet de grand oral soit véritablement républicain ?

dès l'école maternelle. C'est donc un signal que nous envoyons à tout le système scolaire. D'ailleurs, ce signal vaut pour les disciplines en tant que telles, mais aussi pour l'ensemble des activités. Je pense à l'éducation artistique et culturelle,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le baccalauréat fait partie de notre paysage depuis plus de deux siècles. Autant dire qu'il constitue désormais une véritable institution, dont chaque famille s'est saisie, d'autant plus saisie, d'autant plus depuis la massification de l'accès à ce diplôme, décrétée au beau milieu des années quatre-vingt. Réformer le baccalauréat, c'est donc s'adresser à chacune de ces familles concernées à

aux professeurs, qui appliquent bon gré mal gré les différentes réformes voulues par les ministres qui se succèdent. Il n'est pas question pour moi de trancher la question

Nous aurons la justice sociale par l'élévation du niveau général, et l'élévation du niveau général par la justice sociale. C'est le sens, par exemple, du dédoublement des classes de CP et de CE1. C'est le sens de la priorité donnée à l'école primaire et de notre volonté que les élèves entrant dans l'enseignement secondaire maîtrisent les savoirs fondamentaux, alors même que, aujourd'hui, vous

conditionné par les observations des acteurs de l'enseignement supérieur, notamment les professeurs d'université et de classes préparatoires, qui nous ont signalé, par exemple en sciences ou dans les disciplines mathématiques que vous évoquez, un affaissement du niveau, probablement lié au fait que les programmes ne sont pas suffisamment approfondis.

avec un objectif que vous avez affirmé, monsieur le ministre : que le lycée devienne réellement un tremplin pour la réussite de tous les élèves. En effet, notre réalité est la suivante : seuls quatre enfants d'ouvriers non qualifiés sur dix aujourd'hui sont bacheliers. Ces écarts sont plus importants encore pour les filières dites « d'excellence » : quelque 41 % des enfants de cadres supérieurs obtiennent un bac S,

J'ai pu le constater ces dernières années, les dispositifs de carte scolaire, les acteurs en charge de leur mise en oeuvre, leur appropriation ou non par les parents peuvent renforcer- peuvent renforcer- ou non -les inégalités sociales face à l'école. J'avais d'ailleurs dressé ce constat dans un rapport de 2012, qui est malheureusement resté sans suite. Alors que les lycées devraient laisser le libre choix de la combinaison des spécialités à l'élève, alors que le recteur sera le garant de la bonne répartition et de l'équilibre des spécialités sur le territoire, alors qu'un premier trimestre doit être dédié à l'accompagnement dans la construction du projet, il est très clair que des politiques de régulation et d'accompagnement sont primordiales. Ma question est la suivante : quel budget et quels outils de régulation le Gouvernement entend-il développer afin d'éviter que certains enfants ne soient défavorisés ou victimes d'un déficit d'information ? La parole est à M. le ministre.

Mme Sonia de la Provôté. Monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la réforme du baccalauréat ne peut être dissociée de la refonte du lycée et- nous y tenons -d'une réforme de l'orientation pour accompagner le jeune au moins depuis le collège jusqu'au lycée, voire après. L'objectif est, pour chacun, la réussite dans la voie choisie et dans la future vie professionnelle. Si l'on considère la question de l'orientation, celle-ci répond à un véritable défi, à un idéal à atteindre : celui du choix éclairé du jeune sur son avenir. Se pose la question des moyens et des outils pour effectuer ce choix. Un jeune acteur de ses choix est capable de mesurer la meilleure option entre ses goûts, ses envies et ses compétences, indépendamment de sa situation sociale, géographique ou familiale. La mise en place de disciplines de spécialités facultatives, en plus d'un tronc commun, renforce la construction de ce choix. Prévoir plus de souplesse et de liberté dans les combinaisons d'enseignement, c'est servir ce projet. Se pose donc tout naturellement la question de l'information sur les filières, les métiers, les parcours et les carrières. Pour Pour qu'un jeune arrivant au lycée à quinze ou à seize ans puisse décider de façon éclairée de ses études, il doit avoir accès à cette information, en lien avec la réalité du monde du travail.

du jeune. Plus il y a une marge de liberté, plus cela profite aux mieux informés. Les déterminismes sociaux pèsent encore lourd sur la réussite des élèves en France. Monsieur le ministre, nous aimerions connaître la méthode, le calendrier, les moyens et les services que vous allez mettre en place afin de garantir au mieux un choix éclairé pour nos lycéens. Réformer le baccalauréat n'a de sens, vous en conviendrez, que si cette organisation existe vite et sans demi-mesure ! La parole est à M. le ministre.

d'équilibre en ce qui concerne la temporalité. Bien entendu, vous avez entièrement raison : l'ensemble de cette logique réclame une évolution de notre système d'orientation, évolution dont nous avions de toutes les façons besoin. Cette évolution est amorcée, mais elle ne sera pleinement mûre qu'au fil de la réforme.

lieu de mémoire de l'identité française », selon Pierre Nora, le baccalauréat a fait l'objet de nombreux débats. Si nous ne sommes pas opposés à une réforme de cet examen, nous ne pouvons qu'exprimer notre vive inquiétude face à l'imprécision de nombreux aspects de ce chantier, dont la mise en oeuvre est lancée. Il existe d'abord des inquiétudes relatives à l'organisation. Les chefs d'établissement n'ont aucune visibilité sur les modalités pratiques pour le moment : difficultés dans l'organisation des emplois du

entraînera des difficultés de transport, d'aménagement d'emplois du temps et de responsabilités ! Ce lycée modulaire, proche du modèle britannique, risque fort d'entraîner une spécialisation des établissements. Dès lors réapparaîtront des filières officieuses. L'élève « entrepreneur » de son parcours choisira dès demain des spécialités : devront-elles nécessairement être en lien avec son futur parcours universitaire, le premier grade universitaire ? Ces choix précoces et pas très éclairés risquent fort de se faire au détriment des élèves venant des familles les plus défavorisées ! Avec 2 600 postes en moins- administratifs et de professeurs -, comment entendez-vous mettre

La parole est à M. Laurent Lafon. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le succès du nouveau bac dépend en partie de la façon dont les établissements vont se l'approprier. Ma question portera donc sur la marge de manoeuvre et sur la liberté d'action qui sera la leur, notamment sur trois sujets concrets : le recrutement, le temps de travail et l'organisation.

pas faire preuve de souplesse pour aider à mettre en place ces deux enseignements ? En matière de temps de travail, les obligations de service des enseignants sont aujourd'hui fixées de manière hebdomadaire. Cette réglementation nationale empêche les chefs d'établissement d'expérimenter des solutions pédagogiques innovantes sur la périodicité des enseignements ou sur la semestrialisation de l'année scolaire. Le temps Le temps n'est-il pas venu d'avancer sur l'annualisation des obligations de service, comme l'ont proposé de nombreux sénateurs- je pense à Gérard Longuet, mais aussi à Max Brisson et à Françoise Laborde. Pour finir, Pour finir, en matière d'organisation, les établissements ont également besoin de souplesse pour s'adapter aux besoins des élèves et aux spécificités des territoires. Vous avez repris la proposition de réseau du rapport de Pierre Mathiot. D'autres propositions- je pense en particulier à la liberté pédagogique dans le dernier trimestre

M. le ministre. Monsieur Grosperrin, je puis non seulement rassurer la communauté éducative, mais même l'enthousiasmer ! J'ai l'habitude de dire, dans les assemblées de proviseurs auxquelles je faisais référence, que cette réforme n'est pas de l'huile de foie de morue, mais de la vitamine C

est à Mme Claudine Lepage. La réforme du baccalauréat concernera bien entendu également les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger. Cette année, le taux de réussite au 117 609 candidats, quelque 17 134 ont été reçus. En tant que parlementaire représentant les Français de l'étranger, je suis très attachée au bilinguisme, voire au plurilinguisme, indispensable dans le monde d'aujourd'hui.

Pourquoi ne pas encore renforcer et développer l'enseignement des langues dans les lycées en France ? L'expérience du réseau AEFE prouve qu'il est parfaitement possible aux élèves d'étudier trois langues sur une même période. ailleurs, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir à quelle date les élèves du réseau AEFE bénéficieront du numéro d'identifiant national élève, ou INE. Ils n'en ont pas actuellement, et cette absence est très dommageable, puisque les élèves de seconde ne pourront pas effectuer le test numérique de positionnement en français et en mathématiques faute de cet identifiant. Dans le cadre des inscriptions au portail Parcoursup, l'absence de cet identifiant est également très préjudiciable. Les familles doivent saisir manuellement tous les bulletins scolaires. Les élèves ne peuvent pas effectuer les démarches de téléinscription à l'université dès le mois de juillet. Ils doivent attendre la fin du mois d'août et leur arrivée en France pour effectuer la démarche d'inscription. Afin de garantir les mêmes droits à ces élèves, il me paraît urgent, monsieur le ministre, de trouver une solution rapide à ces difficultés d'ordre technique. La parole est à M. le ministre.

qui permettra la prise en compte d'une partie des notes dans Parcoursup et mettra un terme à un mois de juin sans cours. C'est le cas du renforcement de l'oral. L'introduction du contrôle continu dans la notation finale, à hauteur de 40 %, aurait pu être également considérée comme un élément positif. Toutefois, ces 40 % seront en fait constitués pour 10 % des notes du livret et pour 30 % de notes issues d'épreuves de type « bacs blancs » ou partiels organisées à partir de sujets tirés d'une banque nationale. Je crains donc que, à l'inverse de l'objectif, nous assistions à un étalement du bachotage tout au long des classes de première et de terminale, puisque, concrètement, les élèves entreront dans des périodes de révisions à répétition, et qu'à défaut de contrôle continu, on ait plutôt du bachotage continu. Cela pourrait également mener à un formatage de ces rendez-vous dans chaque établissement. Ils rythmeront leur cadre pédagogique et empêcheront ainsi les initiatives plus innovantes, qui ne peuvent reposer que sur la liberté donnée aux enseignants. Le risque est donc grand que le lycée reste le parent pauvre de l'innovation pédagogique et que le baccalauréat continue de formater la pédagogie. Ma question est donc la suivante.

et ne garantissant pas la réussite dans l'enseignement supérieur : tout plaidait pour une réforme de grande ampleur. La réforme que vous proposez à l'horizon de 2021 peut être un atout pour nos jeunes. La nouvelle organisation des études appelle toutefois l'élaboration de nouveaux programmes d'enseignement. C'est la raison pour laquelle vous avez saisi le Conseil supérieur des programmes, qui a d'ores et déjà constitué une quarantaine de groupes d'experts ayant pour mission de concevoir des projets pour les quatre-vingt-deux nouveaux programmes prévus pour le futur lycée. Il s'agit d'une procédure longue, d'autant plus que les enseignements traditionnels vont être modifiés en profondeur, que la fin des séries générales bouleversera le contenu des matières et que de nouveaux enseignements verront également le jour. Je renouvelle mon soutien à la présidente du CSP, Souâd Ayada, mais j'espère que les tensions internes ne ralentiront pas le rétroplanning de ces programmes. Car, pour les éditeurs de livres scolaires, une véritable course contre la montre est engagée. Nul n'ignore en effet la place du livre scolaire lors d'une réforme d'ampleur ; il constitue le premier outil de mise en oeuvre opérationnelle de cette réforme, auquel les enseignants se réfèrent prioritairement par rapport au Avec la Avec la décentralisation, il ne m'a pas échappé que les régions sont en première ligne pour financer les manuels scolaires papier au lycée. En 2019, il leur faudra intégrer le coût de la réforme sur deux niveaux, seconde et première, pour la voie générale et technologique et sur un niveau pour la voie professionnelle. Selon les estimations de Régions de France, le coût total de la réforme pour un équipement complet des élèves des voies générale et technologique sur deux ans et trois niveaux s'élèvera à plus de 300 millions d'euros. À titre d'exemple, la région Île-de-France devra débourser 30 millions d'euros. Nous leur devons, bien entendu, une visibilité totale à court terme, afin qu'elles déterminent aussi exactement que possible leur politique de soutien en la matière. Je crois savoir que les éditeurs sont en contact avec chacune des régions et sont prêts à fournir conjointement des manuels papier et/ou numériques. Ma question sera précise, monsieur le ministre : à quelle date les programmes définitifs seront-ils publiés, et ce calendrier permettra-t-il à tous les partenaires de l'éducation nationale- enseignants, familles, libraires, régions -de disposer, dès la rentrée de 2019, des nouveaux manuels et ressources pédagogiques ? La parole

Si je reculais devant les organisations syndicales ou les lobbies à chaque occasion, cela se verrait et cela se saurait, et nous ne serions même pas là pour parler de la réforme du baccalauréat ! C'est clairement en fonction de choix

du profil de chaque élève à la formation proposée dans notre système éducatif, et plus particulièrement au baccalauréat. Si la réforme du baccalauréat, que nous appelions tous de nos voeux, va dans le sens d'une meilleure adaptation

Nous connaissons tous la pression sociale qui tend à faire passer le baccalauréat au plus grand nombre d'élèves, comme si ce seul diplôme était à même de garantir la réussite dans le monde professionnel. Pourtant, cette généralisation du baccalauréat, cette fameuse politique des « 80 % de bacheliers », lui a fait perdre son statut et a eu pour conséquence majeure une dégradation de sa valeur. Malheureusement, malgré quelques efforts entrepris, les autres voies scolaires- les filières technologiques ou professionnelles -souffrent d'une image qui va encore trop à l'encontre de l'idée d'excellence académique. Or chacun s'accorde à reconnaître que seule la volonté politique d'un bac plus sélectif serait à même de lui rendre sa vocation première et de permettre à d'autres filières de se développer et de devenir attractives aux yeux des élèves. on accuse chaque année le système de correction du baccalauréat d'être partiellement responsable de la démonétisation de cet examen, les professeurs étant amenés à donner des notes acceptables à des copies qu'ils trouvent pourtant bien en deçà des exigences attendues. Il ne se Il ne se passe plus désormais une année sans que l'on fasse état de dysfonctionnements graves lors des épreuves, de tricheries plus ou moins importantes ou bien de problèmes de notation des candidats. Comme le déplorait un professeur, « décidément, le bac n'est plus un examen équitable ». Ou, comme le dit si bien Michel Fize, dans son livre, « les bacheliers sont de grands bernés de la République est un diplôme coûteux pour la Nation, que de plus en plus d'entreprises recrutent sans, mais sur des tests psychotechniques, et que dans certains pays émergents il n'y a ni notes, ni évaluation, ni diplôme ; et pourtant, à dix-huit ans, les jeunes y sont admis dans les plus hautes écoles supérieures et réussissent fort bien.

Inévitablement, quelques esprits anciens auront la nostalgie de cette épreuve jadis tant redoutée. Comme s'il y avait eu un âge d'or, le temps pas si lointain où bien peu de nos concitoyens pouvaient accéder à cette acropole lycéenne Parce que ses taux de réussite sont désormais particulièrement élevés- près de 90 % -, parce que le nombre de mentions « Très bien » atteint des niveaux records, certains estiment que le baccalauréat est quasiment donné. Ce discours est difficile à admettre pour les néo-bacheliers qui ont travaillé avec coeur et abnégation durant toute l'année pour obtenir ce diplôme. Cependant, il est vrai que l'harmonisation de la notation, dont de nombreux correcteurs ont souvent déploré l'indulgence ou la bienveillance, par son opacité, pour ne pas dire son obscurité, suscite de légitimes interrogations. Régulièrement, de mini-scandales éclatent, pointant les consignes de correction à la hausse émanant des inspecteurs de l'éducation nationale. Pour évacuer cette suspicion de « bac au rabais », et même si l'introduction du contrôle continu va logiquement changer la donne, il serait souhaitable de rendre publics les barèmes de notation. Voilà dix ans, l'un de nos prédécesseurs, le sénateur Jacques Legendre, dans un rapport sur le sujet, regrettait cette absence de transparence autour du processus d'harmonisation. À propos de ces fameuses commissions et des consignes qui y sont données, il écrivait ainsi À tort ou à raison, elles sont soupçonnées de contribuer à augmenter de manière artificielle les taux de réussite et d'affaiblir ainsi la valeur du baccalauréat. » Monsieur le ministre, vous qui êtes un grand promoteur des évaluations dès les plus petites classes, afin d'obtenir une vision objective du niveau des élèves français, allez-vous appliquer cette même ligne de conduite et une volonté de clarté dans la notation pour le nouveau baccalauréat ?

Il est exact qu'il peut se produire parfois des « phénomènes ascensionnels », qui n'ont jamais recueilli pleinement mon assentiment, et que nous devons revenir à une certaine raison en la matière.

Nous sommes parfois un peu frustrés de ne pas pouvoir développer notre raisonnement, et vous-même l'êtes sans doute de ne pas avoir pu répondre dans le détail à l'ensemble des questions qui étaient posées. Vous avez réaffirmé la nécessité que le baccalauréat soit un tremplin pour l'enseignement supérieur. Au Sénat, nous souhaitons qu'il soit, plus largement, un tremplin pour la réussite et l'épanouissement des élèves, ainsi que pour leur insertion professionnelle. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Quel que soit notre territoire, que l'on soit issu des grandes villes, du milieu rural, d'un pays étranger- je remercie Claudine Lepage d'avoir

il nous paraît important que l'équité de cette épreuve soit assurée. Vous l'avez compris, l'équité territoriale est le maître mot ici, au Sénat. Nous voulons donc que soient réunies les conditions de la réussite de cet examen dans sa nouvelle formule.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

en 2011 sur la réindustrialisation, nous avons effectué un travail important tant sur Alstom que sur le redéploiement de notre industrie. Pour cette

et une concurrence exacerbée au niveau international. Comment se fait-il que la France, qui était le premier pays exportateur, avec près de

dire aux parlementaires et aux Européens que nous devons faire en sorte d'être mieux défendus. On ne peut pas demander à nos industriels de s'adapter aux lois

Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire en introduction. Pendant six mois, nous avons travaillé avec une vingtaine de sénateurs et sénatrices à nos côtés.

un accord avec Siemens, mais à égalité, comme dans le cas d'Airbus : deux États, deux groupes et l'égalité entre eux. Pourquoi avoir fait passer un groupe comme Alstom sous la maîtrise allemande ?

Il faut que la France croie de nouveau en son industrie, pour ne pas aller vers le modèle décrit par Michel Houellebecq d'une France vidée de ses usines et ses ouvriers, d'un pays touristique où ne subsisteraient que des stations de ski et des hôtels de charme. charme. La forte désindustrialisation que nous connaissons n'est pas une fatalité. Les propositions que nous présentons nous offrent la possibilité d'avoir un débat avec le Gouvernement, pour essayer de redresser la barre. ce renouveau industriel que nous appelons de nos voeux, avec des propositions concrètes tant sur le financement que sur les politiques de suramortissement qui avaient été votées dans cette assemblée, à l'unanimité, l'année dernière, pour donner à nos PME-PMI la possibilité d'investir dans l'industrie du futur. Il faut favoriser le territoire français

monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de cette invitation à débattre d'un sujet qui me tient à coeur. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de vos conclusions et de vos propositions. Je partage votre sentiment d'urgence, qui s'exprime en particulier dans le second tome de votre rapport. On peut certes se réjouir d'un retour relatif de l'industrie en France en 2017, avec des créations d'emplois, de l'investissement étranger et des ouvertures de sites industriels plus nombreuses que les fermetures, nous sommes bien conscients que les efforts qui restent à mener sont considérables. Nous partageons la même volonté de faire revivre puissamment la France industrielle. Le sursaut doit être accompagné, soutenu et attisé. notre industrie est à la fois notre héritage et ce qui construira notre futur. C'est à la fois la conquête de marchés étrangers et la vitalité économique de centaines de territoires français, notamment ruraux. C'est à la fois notre compétitivité et ce qui garantit notre souveraineté. Cet horizon est vraiment ce qui nous a conduits à engager une transformation en profondeur de notre économie depuis le premier jour du quinquennat, avec un travail en profondeur sur la compétitivité de nos entreprises.

À cela se sont ajoutées les dispositions de la loi Travail pour constituer les deux piliers très puissants de notre politique visant à restaurer la compétitivité de notre économie et de notre appareil productif.

deuxième objectif est de faire de la France la première nation en matière d'innovation en Europe. Cela passe par un investissement massif dans les compétences, dans la recherche et dans notre appareil productif. Notre ambition en la matière se traduit par une politique d'innovation ambitieuse, d'une dimension nouvelle, couplée avec une réforme sans précédent de la formation professionnelle et de l'apprentissage. recherche, le CIR, que vous avez citée, l'État entend jouer pleinement son rôle de stratège et de catalyseur, par des choix d'investissements sur les technologies de rupture avec la création du fonds pour l'innovation et l'industrie, doté doté de 10 milliards d'euros. Ce fonds a commencé à fonctionner, avec deux premiers défis qui portent sur l'amélioration des diagnostics médicaux par l'intelligence artificielle et la sécurisation des systèmes ayant recours à l'intelligence artificielle. Le rôle de l'État n'est pas d'immobiliser des capitaux dans des entreprises lorsqu'il dispose d'autres leviers suffisamment puissants. Il n'a donc pas besoin du contrôle actionnarial pour garantir la préservation des intérêts nationaux. Son rôle est de préparer l'avenir du pays et non pas d'agir en gestionnaire financier. C'est pour cette raison que nous ne donnerons pas un avis favorable à la proposition n° 31 de votre mission d'information. Le deuxième levier pour mettre l'industrie française à la pointe est un travail partenarial conduit entre le Gouvernement et seize filières structurantes pour notre industrie. Je prendrai l'exemple de la filière automobile, qui mobilise l'ensemble des acteurs pour accélérer le développement des véhicules hybrides, électriques et autonomes, ainsi que des nouveaux usages de la mobilité. L'association entre les pouvoirs publics et l'industrie automobile est incontournable si nous voulons le meilleur cadre fiscal, réglementaire et territorial pour mettre notre industrie à la pointe. l'exemple de la filière santé, avec laquelle nous avons bâti un plan d'action complet en juillet dernier, pour réduire les délais d'autorisation des essais cliniques et d'autorisation de mise sur le marché des médicaments et pour préparer les innovations de demain, la création d'une plateforme de partage des données de santé qui sera sans doute l'une des plus riches du monde. Enfin, nous voulons ancrer nos outils de soutien à l'innovation dans les territoires. J'ai ainsi lancé en juillet dernier un appel à candidatures pour « relabelliser » les pôles de compétitivité et lancer une phase 4 d'ambition européenne. nous ne sommes pas naïfs : la préservation de notre autonomie dans certaines technologies stratégiques est indispensable pour garantir notre souveraineté économique. Nous devons pouvoir rester maîtres de nos innovations. Car à quoi bon investir dans les technologies de rupture si c'est pour se faire piller ses investissements quelques années plus tard ? Dans la loi PACTE, nous renforçons le régime de contrôle des investissements étrangers en France, en élargissant le champ du contrôle à de nouveaux domaines, notamment l'espace, le stockage de données, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Sur ce point, les propositions de votre mission sont pleinement en accord avec notre vision. vision. Sur ce sujet de la souveraineté économique, j'aimerais évoquer la fusion entre Alstom et Siemens. C'est pour préserver une souveraineté économique européenne face à un géant industriel chinois que cette fusion a été décidée. Le rapport de votre mission a conclu que la fusion actuelle était la meilleure option pour faire naître un géant européen du ferroviaire, même si j'ai bien entendu que vous en contestiez les modalités financières et capitalistiques. Mais il était vital Mais il était vital d'aboutir sur ce rapprochement et tout aussi crucial de défendre les intérêts français. Une série d'engagements ont été pris pour fixer le siège de la nouvelle société et sa cotation en bourse en France, ainsi que pour assurer l'équilibre de sa gouvernance. Siemens s'est également engagé à préserver le niveau d'emplois pendant quatre années. Il s'agit ainsi d'un mariage entre égaux, mais avec une situation actionnariale asymétrique que vous avez déplorée. L'État veillera à ce que l'équilibre entre la France et l'Allemagne perdure. Vous avez également évoqué dans le rapport de votre mission des points de vigilance, en particulier sur la sous-traitance et l'animation de la filière. Je vous rejoins sur ces points et serai attentive à ce que les engagements pris soient tenus. La nouvelle entreprise devra continuer à développer un socle de fournisseurs solide en France et en Allemagne. S'agissant des commandes pour les marchés français et allemand, elle devra recourir préférentiellement aux fournisseurs du pays. Plus généralement, notre politique industrielle ne peut rester cantonnée aux grands groupes et aux grandes métropoles. Une bonne politique d'innovation dans l'industrie doit entraîner toutes les PME, dans tous les territoires. C'est pourquoi nous faisons porter l'effort principalement sur les PME, avec une nouvelle grande étape de réformes structurelles, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Notre premier défi est de consolider l'ensemble de notre appareil productif, car notre tissu économique est trop fragile. Nos entreprises rencontrent des obstacles accumulés dans des strates réglementaires et fiscales qui les freinent à toutes les étapes de leur développement. Elles sont donc trop petites et mal financées ; elles n'innovent et n'exportent pas assez. Nous allons faciliter la création, le financement, la transmission et le rebond des entreprises. Le deuxième défi est celui de la transformation numérique de notre industrie : le Gouvernement est pleinement engagé pour combler le retard qu'a pris la France dans la digitalisation et la robotisation de son industrie. Les annonces faites par le Premier ministre il y a quelques jours concernant l'industrie du futur et l'ensemble des mesures de soutien à la modernisation et à la numérisation de nos entreprises sont absolument cruciales

dans chacune des filières du Conseil national de l'industrie, d'une plateforme numérique pour accompagner à la numérisation, filière par filière. Enfin, une mission sur les plateformes d'accélération de l'industrie du futur a été lancée. consiste à ancrer notre politique industrielle dans chaque territoire. C'est ce que nous faisons au travers de l'initiative « Territoires d'industrie », portée par les ministères de l'économie et de la cohésion des territoires.

Pour conclure, les 45 propositions de la mission d'information en matière de stratégie industrielle pointent, pour une grande majorité, dans la même direction que les actions entreprises par le Gouvernement. Je veux saluer encore une fois la qualité de l'analyse que vous avez menée et me féliciter du débat que nous allons avoir aujourd'hui. Nombreuses sont les recommandations qui vont trouver leur place dans la loi PACTE, notamment sur l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés, sur le développement de l'épargne salariale ou sur le renforcement du décret sur les investissements étrangers en France.

à renouveler sa stratégie industrielle. Mais si nous considérons que la dynamisation de l'outil actionnarial peut être un levier possible pour servir cette nouvelle stratégie d'État,

sera médiocre pour financer le soutien de l'innovation de rupture qui fera l'économie de demain. Contrairement à ce qui a été dit au départ, et que vous avez répété à l'instant, madame la secrétaire d'État, ce ne sont pas 10 milliards d'euros qui vont être affectés à ce soutien, mais le produit des dividendes engendrés par le placement des actions que vous allez vendre. Comment justifiez-vous que les placements de ces 10 milliards d'euros produiront un rendement de 250 millions d'euros au mieux, alors que, aujourd'hui, et en prenant appui sur les chiffres des années passées, les actions de ces trois entreprises ont rapporté à l'État 850 millions d'euros au plus bas en 2017 et jusqu'à 1,5 milliard d'euros les

pour l'État ? Certes, vous allez réintégrer immédiatement 10 milliards d'euros qui vous éviteront peut-être de passer en 2019 le cap symbolique des 100 % de PIB de dette publique, mais quelle est la véritable logique de cette opération de vente et d'abandon de fleurons nationaux ?

de faire de l'État un État stratège, plutôt qu'un État gestionnaire ou rentier. Nous préférons investir dans les technologies de demain, plutôt que de rester actionnaires dans des entreprises qui, certes, produisent un rendement,

ces cessions d'actifs seront réalisées dans un cadre extrêmement sécurisé du point de vue de la régulation. Il s'agit effectivement d'un choix d'allocation de l'argent public vers d'autres priorités. Encore une fois, ce choix d'un placement en obligations d'État, donc d'un rendement

Pour éviter de revivre la calamiteuse opération des autoroutes de 2005, il faut que le produit des ventes de ces trois entreprises soit au moins égal à la somme actualisée sur très longue période du produit des dividendes auquel l'État va renoncer. C'est ce que nous examinerons avec attention, mais nous espérons que vous saurez éventuellement arrêter le processus de privatisation si vous ne pouviez parvenir à préserver les intérêts de l'État et des clients de ces entreprises- c'est aussi un sujet en soi -, mais aussi ceux des propriétaires, les Français.

Dans ma région des Hauts-de-France, nombre d'industries, de l'automobile au textile, en passant par la métallurgie, ont mis la clé sous la porte. Entre 2017 et 2018, le Nord-Pas-de-Calais a encore perdu 1 400 emplois industriels ; en dix ans, ce chiffre atteint plus de 70 000 emplois. industries qui subsistent connaissent des difficultés ou font état de grandes inquiétudes sur leur avenir. Je citerai plusieurs exemples pour illustrer mon propos. L'entreprise Balsan, située à Calais, est spécialisée dans la fabrication des tenues des grands corps militaires, tels que la Garde républicaine ou l'École polytechnique. Surtout, l'entreprise est titulaire du marché de l'Armée de terre. Elle détient un savoir-faire unique dont la valorisation n'est pas prise en compte dans les procédures de passation des marchés. Il existe donc un risque fort de bascule de ce marché vers une entreprise étrangère. Lors d'une dernière répétition du défilé du 14 Juillet, le général François Lecointre en montant dans le véhicule présidentiel : l'entreprise calaisienne l'a remplacée en moins de vingt-quatre heures. Deuxième exemple récent, la perte de marché de Protecop au profit d'une entreprise irlandaise n'est pas pour nous rassurer. Là où dix sous-traitants français auraient pu vivre d'un marché de 300 000 gilets pare-balles- c'est d'actualité -, l'Irlandais assure sa production en Asie. Que dire de la situation d'Ascoval, à Saint-Saulve, aciérie de près de 300 salariés qui est en redressement judiciaire depuis janvier Deux repreneurs se sont positionnés, mais l'actionnaire principal, Vallourec, propose un tarif d'achat de l'acier produit très inférieur au prix du marché et insuffisant pour garantir le modèle économique d'Ascoval. Or l'État détient 16 % du capital de Vallourec ; il est donc en mesure de peser dans les négociations.

circulent. Aussi, j'aimerais connaître quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour respecter l'engagement du Président de la République de maintenir une industrie forte et compétitive pour notre pays, afin que nos salariés puissent, selon la formule qu'il avait employée lors de sa visite sur le site d'Ascoval, « dormir sur leurs deux oreilles ». La parole est à Mme la secrétaire d'État.

positionnées respectivement sur les uniformes et les équipements de protection individuelle. Je salue la transformation qu'elles ont su apporter, l'une et l'autre, à leur offre, avec un service sur mesure

une mauvaise nouvelle. La direction des achats de l'État du ministère de l'économie et des finances échange de manière permanente avec les ministères concernés et veille à ce que, même dans un contexte budgétaire contraint, les modalités de choix des fournisseurs tiennent compte au mieux des qualités et spécificités des produits des entreprises concernées et maximisent le recours aux entreprises nationales. Le contexte juridique est néanmoins contraint par les règles des marchés publics et les règles européennes en la matière. S'agissant de l'entreprise Ascoval, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir à l'occasion d'une autre question, que les services de mon ministère sont extrêmement présents sur ce dossier. Leur rôle est d'accompagner les propositions de reprise, pour s'assurer qu'elles sont solides et crédibles. C'est bien la phase dans laquelle nous sommes actuellement, avec des projets de reprise qui doivent encore être travaillés,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, l'avenir de notre industrie automobile dépendra de sa capacité à innover et à s'adapter au développement du véhicule électrique, mais aussi à prendre en compte les enjeux du développement durable. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, je vous interroge sur le bouleversement qui s'annonce et qui sera tout aussi radical que le passage de la machine à vapeur au moteur à explosion. Je me réjouis de constater que le véhicule électrique va prendre toute sa place, avec une part de marché qui va bondir de 1 % à 30 % d'ici à 2030. Autant dire que les constructeurs, mais également les garagistes, les équipementiers et les pétroliers vont affronter un véritable, une une révolution importante pour répondre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la diminution de la dépendance énergétique au pétrole du secteur des transports et à l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain.

Si les véhicules électriques sont propres, leur fabrication, avec les matériaux qui composent les imposantes batteries et les métaux rares de la partie électronique, ne l'est pas vraiment. En effet, les batteries au lithium des voitures électriques contiennent des matériaux polluants, ce qui implique de proposer leur recyclage, dans le cadre de la protection de l'environnement. Pour que la voiture électrique soit vraiment intéressante sur le plan environnemental, il est primordial de mettre en place des filières de recyclage des batteries. Aussi, dans le cadre de la mission d'information que j'ai présidée en 2016 sur le devenir des composants des téléphones mobiles, il a été souligné l'insuffisance de la collecte des téléphones inutilisés, puisque 100 millions de téléphones dorment dans les tiroirs des Français. Seuls 15 % des téléphones portables usagés sont collectés. C'est pourquoi la mission a effectué plusieurs propositions visant à mettre en oeuvre une stratégie nationale de recyclage des métaux, en s'inspirant des deux déplacements effectués auprès d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans les Deux-Sèvres et d'un site industriel de recyclage des métaux précieux à Anvers.

est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur Longeot, vous avez absolument raison : nous avons bien identifié le recyclage des batteries comme un enjeu majeur pour le développement de la mobilité électrique. batteries de la mobilité sont notamment constituées de ressources rares- le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares -, peu ou pas produites en Europe. Les compétences françaises existent, en revanche, dans la R&D et la mise en oeuvre du recyclage des batteries. La France est active,

Des compétences industrielles nationales existent dans la récupération de métaux critiques, et des compétences de recherche de haut niveau dans la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Des projets stratégiques sont en cours de définition, notamment dans le cadre du comité stratégique de filière « Mines et métallurgie » du Conseil national de l'industrie. En effet, celui-ci a inscrit dans son contrat de filière le projet structurant de développement d'une filière intégrée du recyclage des batteries lithium. L'enjeu est de faire émerger en France une filière leader dans le recyclage des batteries, utilisant les meilleures technologies disponibles et s'appuyant sur un modèle économiquement soutenable. Le Gouvernement examine avec intérêt ce projet et soutient la filière de recyclage des batteries de véhicules électriques, tant en amont, dans la R&D, qu'en aval, dans l'accompagnement de l'émergence d'un industriel spécialisé et performant.

Force est de constater que, depuis quelque temps, la France a perdu une part de sa souveraineté. En effet, avec Alstom, elle a cédé ses turbines et ses réseaux électriques, après avoir vendu ses téléviseurs, son imagerie médicale, son aluminium, son acier et son ciment,

comme l'est le conglomérat américain pour la branche énergie. La vérité est que nous assistons à une braderie des intérêts stratégiques français au profit d'intérêts étrangers. Nous avons donc manqué l'occasion de créer un Airbus du rail, un groupe fondé sur une relation équilibrée, gagnant-gagnant, qui préserve les savoir-faire, les technologies et les emplois. Rappelons que General Electric avait promis de créer 1 000 emplois. Où sont-ils ? Avons-nous donc, par le choix malheureux de Siemens, perdu la bataille du rail

en particulier pour Aéroports de Paris et la Française des jeux, une régulation renforcée, extrêmement précise et surtout protectrice du consommateur.

Pour autant, l'intervention capitalistique de l'État doit s'effectuer avec parcimonie, au regard de la situation des finances publiques et aussi des règles européennes. C'est pourquoi notre mission a estimé qu'il pouvait être souhaitable de redéfinir le niveau des participations de l'État dans certaines entreprises, sans tabou de principe, pour les recentrer, le cas échéant, sur les actifs les plus stratégiques.

de mes collègues dans cet hémicycle ... En outre, toute réorganisation ou réorientation de l'actionnariat de l'État, qui conduirait notamment à faire perdre à ce dernier la qualité d'actionnaire majoritaire ou d'actionnaire de référence d'une entreprise stratégique, doit intervenir parallèlement à la mise en place de mécanismes d'information, de contrôle et de décision spécifiques, afin qu'il garde des moyens d'action lorsque les intérêts de la Nation sont en jeu. Cela est particulièrement vrai à l'heure où le projet de loi PACTE organise les conditions de la cession des participations de D'autre part, il nous semble que les sommes découlant de ces cessions d'actifs ne doivent pas être uniquement réservées au fonds pour l'innovation de rupture ou aux start-up. Il faut pouvoir réinvestir directement dans certaines entreprises aux activités plus classiques,

avant que certaines décisions lourdes de cession ou d'investissement ne soient prises. Sur ces différents points, je souhaiterais vous entendre.

très fermes de régulation, d'information et de droit de regard de l'État sur un certain nombre de décisions qui concernent ces entreprises. J'ajoute que le projet de loi PACTE comporte aussi une modernisation des dispositifs d'action spécifique,

le portefeuille d'actionnariat de l'État est quelque chose de vivant, qui doit être géré avec agilité ; or il me semble que M. Chatillon, qui représente le Sénat en matière de participations de l'État, n'est pas suffisamment informé au fil du temps. Il faut donc prévoir un dispositif d'association du Parlement

avec des gammes de produits un peu démodés, un peu anciens ; nous sommes peu présents à l'exportation ; notre compétitivité est faible. Il y a donc une action importante à mener.

vous avez raison : nous avons certes besoin de leviers dans différentes dimensions, encore faut-il que tous ces leviers s'appuient les uns les autres. Il faut aussi que nous sachions travailler avec les régions. De plus en plus, les partenariats avec les régions sont indispensables pour faire avancer

à la fois par filière et par thématiques transversales, numérique et export, qui nous donne cette approche matricielle et qui fait tenir ensemble les différentes dimensions de notre politique industrielle. Les marchés publics aux États-Unis ? Ce n'est pas un sujet facile. Nous disposons

Je ne vous cache pas que ce dossier est complexe à faire avancer. Enfin, la politique industrielle européenne est l'un des grands sujets que nous voulons porter à l'agenda de la prochaine Commission. Nous avons commencé à y travailler avec nos partenaires européens, en échangeant des papiers de problématique et en cherchant

d'un secteur industriel considéré comme stratégique par l'État français. Le besoin de transport est une réalité toujours plus importante, en France et en Europe. Le transport ferroviaire est l'une des réponses aux défis de l'aménagement du territoire et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les contrats de commande publique signés par Alstom sont énormes.

et sur les sous-traitants auxquels l'entreprise fera appel. Cela a déjà des conséquences. Par exemple, un sous-traitant métallurgique a déjà fait faillite cet été près de La Rochelle. Par ailleurs, Alstom pousse toujours l'externalisation vers des pays socialement moins-disants- j'aurais beaucoup à dire sur l'usine de Katowice. Autre exemple : l'usine de Belfort. Le contrat pour vingt-deux locomotives de manoeuvre, dont la SNCF a besoin, ne lui est toujours pas attribué, et Alstom n'investit plus dans cette usine. réponse à la question de l'avenir industriel de notre pays passe par le traitement de ces questions concrètes, celles du lien entre commande publique et stratégies de conception et de production en France et en Europe. L'absorption d'Alstom par Siemens ne semble pas remise en cause par l'État, alors qu'elle l'est par l'autorité de la concurrence européenne et même par les autorités britannique et australienne ! Ce qui est pire, l'État français continue de préciser qu'il n'entrera pas au capital de la société, alors même qu'il avait des droits de vote chez Alstom et que Bouygues veut en sortir. Madame la secrétaire d'État, il semble que les mêmes erreurs se répètent. Comment pouvez-vous encore justifier une telle absorption d'Alstom par Siemens ? Pourquoi les questions des salariés et des syndicats d'Alstom

ferroviaire, nous nous attachons à faire en sorte que le carnet de commandes du donneur d'ordre profite à l'ensemble de son écosystème d'entreprises en France. C'est d'ailleurs aussi l'esprit des accords que nous avons passés au moment du rapprochement avec Siemens.

commandés par la SNCF fin juillet. Lors de sa venue dans les Hautes-Pyrénées en juillet dernier, le PDG du groupe Alstom m'a confirmé ses propos tenus lors de son audition par la commission des affaires économiques : le d'Alstom à Tarbes étant considéré comme un centre de compétence mondial en matière de recherche et développement, et donc comme moins susceptible de subir des creux de charge, son avenir ne semble pas compromis. Au vu des récentes commandes, nous avons toutes les raisons de le croire. En effet, le site tarbais est l'un des fleurons de notre industrie, et il est capital de maintenir ce bassin d'emplois vital pour notre pour notre territoire- mais jusqu'à quand sera-ce possible ? Cela étant dit, la direction a soulevé, lors de sa visite, la question importante de la commande publique en France. La commande des trains à hydrogène est un exemple parlant : c'est l'Allemagne qui fait cette commande. C'est une bonne nouvelle pour l'usine de Tarbes. ailleurs, la région Occitanie est l'un des principaux clients du site pyrénéen. Ne faudrait-il pas, dès lors, encourager les régions, mais aussi des opérateurs comme la SNCF, à diversifier leurs projets et à oser des expérimentations telles que le train à hydrogène pour dynamiser les sites de production français ? Madame la secrétaire d'État, quelle stratégie comptez-vous mettre en oeuvre pour favoriser et développer le maintien de la commande publique aux entreprises industrielles françaises et pérenniser nos sites de production en France ?

est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous évoquez le cas du site de Tarbes et de la technologie hydrogène pour le ferroviaire. Nous avons tous, en effet, été frappés par l'annonce

décarbonée est l'un des axes sur lesquels nous travaillons. Plus généralement, pour toutes celles et tous ceux qui ont des questions relatives à des sites ou à des territoires en particulier,

volonté est donc de préserver l'outil industriel et sa capacité d'innovation et d'investissement, ainsi que les compétences associées. Encore une fois, je suis persuadée que l'excellence des sites français et des ingénieurs et chercheurs français

sujet ! La parole est à Mme Valérie Létard. Je suis particulièrement attentive à l'évolution du secteur industriel dans notre pays. Dans ma région, les Hauts-de-France, l'industrie emploie aujourd'hui plus de 300 000 personnes. Le secteur industriel y est en mutation permanente. Nous pouvons nous réjouir de bonnes nouvelles, comme les investissements engagés par Toyota ou encore les commandes passées au site Alstom de Petite-Forêt pour le Grand Paris Express. Encore faut-il qu'Alstom poursuive poursuive la modernisation de cette usine en engageant les investissements attendus et rassure ainsi sur la pérennité, à terme, de ce site d'excellence, ainsi que sur sa volonté de recourir à des sous-traitants nationaux. D'autres secteurs rencontrent des difficultés- je pense en particulier à l'aciérie Ascoval, qui appartenait au groupe Vallourec. Le 29 juin 2015, le ministre Emmanuel Macron, en visite sur le site de l'aciérie Ascoval, déclarait : « Il s'agit d'une aciérie qui est au plus haut niveau de qualité et de qualification. Le 22 janvier dernier, le Président Macron, en visite chez Toyota, a eu des paroles rassurantes en direction de la maire de Saint-Saulve, Cécile Gallez, sur l'avenir d'Ascoval, alors en procédure de redressement judiciaire. Aujourd'hui, comme vous le savez, un repreneur, Altifort, a déposé une offre sérieuse pour reprendre Ascoval. Robuste d'un point de vue industriel, commercial et économique, selon le cabinet Secafi, le projet d'Altifort consiste à installer un nouvel outil : un train à fil. Altifort reprendrait les 281 salariés actuels au démarrage du nouvel outil ; l'emploi passerait à terme à 414 salariés. Mais Altifort a besoin du support de Vallourec pendant une période de dix-huit mois, le temps de construire et de démarrer le train à fil. Il s'agit d'obtenir de Vallourec l'engagement de maintenir un volume d'activité aux conditions actuelles, et pas davantage. Le 25 septembre dernier, le ministre Bruno Le Maire a réuni la direction et les représentants des salariés d'Ascoval. En conclusion de cette réunion, le ministre a indiqué que l'ensemble des acteurs devait travailler de manière exclusive à ce scénario de reprise auquel il croyait. Enfin, il a indiqué que l'État se chargeait de la négociation avec Vallourec, Alors que l'offre d'Altifort doit être remise le 19 octobre prochain, pouvez-vous nous faire un point sur les négociations que le Gouvernement s'est engagé à mener avec Vallourec ?

et de présenter une perspective crédible à l'entreprise et aux salariés. Nous souhaitons vraiment mesurer les points forts et les faiblesses des projets de reprise soumis au tribunal. Nous savons que le secteur de la sidérurgie est particulièrement complexe avec des retournements de conjoncture et un environnement international qui peut être instable, voire créer des difficultés temporaires assez aiguës. Le Maire, la semaine dernière, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé un délai supplémentaire de quatre semaines afin de permettre aux divers repreneurs potentiels de finaliser leur projet pour Ascoval. Il existe aujourd'hui deux projets, et nous sommes en contact avec les deux repreneurs. Aucun d'eux ne semble disposer, à ce stade, des financements importants indispensables ; le sursis accordé par le tribunal leur permet d'essayer de les rassembler.

Encore une fois, nous déployons toute l'énergie possible pour trouver une solution viable dans le dossier Ascoval. C'est compliqué, les salariés en sont conscients. Nous y travaillons de façon extrêmement sérieuse et assidue. La parole

de disposer d'une véritable visibilité industrielle dans la planification des besoins et la programmation des projets ferroviaires. Il en va de même pour d'autres projets d'investissement dans notre pays. Réduire les effets cycliques, qui fragilisent les donneurs d'ordre et les fournisseurs de cette industrie, est évidemment une priorité. En France, comme ailleurs, la puissance publique- les agglomérations, les régions, l'État -est au coeur de l'écosystème et arbitre les modalités de la commande publique. La filière industrielle ferroviaire doit pouvoir compter sur une visibilité à quatre ou cinq ans afin de mieux anticiper les besoins et d'organiser son outil son outil industriel. Madame la secrétaire d'État, quelles initiatives de programmation pourraient être mises en place pour soutenir des activités importantes pour nos territoires ?

Dans un contexte fortement concurrentiel, le prix devient de plus en plus l'unique facteur d'attribution des marchés. Nous connaissons tous certains enjeux du commerce international et la réalité des coûts horaires variables suivant les lieux de production. Pour les offres françaises, il serait donc opportun de réfléchir à la valorisation de critères techniques et de clauses RSE soutenant l'ancrage d'activités en France. L'exigence de compétitivité des projets est assurément indispensable indispensable et normalement génératrice d'une saine émulation. Il ne faudrait pas que cet objectif s'oriente systématiquement vers un choix du « moins-disant » en termes de prix. L'industrie française n'y résisterait pas. Nos emplois, nos compétences, la vitalité de nos territoires sont en jeu. La France et, plus largement, l'Europe doivent pouvoir s'engager dans ces démarches responsables. Comment le Gouvernement entend-il soutenir avec d'autres parties prenantes cette nouvelle approche ? La parole est à Mme la secrétaire d'État.

La Haute-Vienne abrite néanmoins diverses unités de production industrielle, souvent de petite taille, mais aux savoir-faire extrêmement pointus. Elles collaborent avec de grandes marques du haut de gamme français, s'inscrivant ainsi totalement dans la démarche de qualité du, même si je préfère, pour respecter notre belle langue, parler du « fabriqué en France ». du « fabriqué en France ». Très bien ! Au-delà de la traditionnelle et réputée production de porcelaine, comment ne pas citer le secteur de l'habillement de luxe ou haut de gamme avec, par exemple, le chausseur Weston et France Confection, à Limoges- cette dernière entreprise fournissant notamment les costumes de haute qualité de la marque Smuggler et de bien d'autres Je pourrais aussi citer les peausseries à Saint-Junien, où Hermès, désireux d'optimiser les savoir-faire locaux, a implanté une unité de production et où existent, depuis longtemps, des fabriques de gants de haute qualité- je pense, entre autres marques, à Morand et Agnelle. Les élégantes chaussettes Archiduchesse et Bonne Maison,

Pour autant, l'installation de ce type d'unités de production et leur maintien en France s'avèrent complexes et incertains. Elles sont souvent fragilisées non seulement par une fiscalité inadéquate, mais aussi, et surtout, par des difficultés de recrutement de main-d'oeuvre. Le maintien d'une politique industrielle territorialisée passe par une meilleure coordination de l'action des pouvoirs publics à l'échelon local. Il passe aussi et surtout par la revalorisation des métiers et des formations industriels, trop peu prisés par la jeunesse. Créer, par exemple, des « classes d'excellence » dans le domaine de l'apprentissage et faire des métiers de l'industrie un axe majeur du plan d'investissement dans les compétences pourrait contribuer à cette nécessaire revalorisation.

-qui sait ce que le mot « désindustrialisation » signifie et combien néfastes peuvent en être les conséquences sur le territoire ; je pense notamment aux crises de la sidérurgie, des mines et du textile.

Sur la scène internationale, la transformation s'est opérée à une vitesse vertigineuse. Elle a conduit à une profonde modification des rapports de force mondiaux

La part des exportations françaises dans le commerce mondial ne cesse de diminuer : la France, deuxième puissance économique de la zone euro, perd encore et toujours des parts de marché à l'exportation. L'importance de l'industrie dans l'économie française ne cesse de décliner.

Notre modèle industriel doit s'adapter aux mutations technologiques, à la robotique et aux enjeux environnementaux. Madame la secrétaire d'État, comment le Gouvernement compte-t-il déployer sa stratégie de reconquête industrielle et commerciale et avec quels moyens financiers, tout en favorisant la qualification et la formation des hommes ? La parole est à Mme la secrétaire est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Husson, il s'agit en effet de mettre un coup d'arrêt à la désindustrialisation et de déployer une stratégie de reconquête. Je reprends vos mots, qui me semblent parfaitement adaptés.

au profit de l'industrie de demain, la mobilisation collective de l'industrie et des filières sur les nouveaux marchés et la transformation numérique de l'industrie à travers la présentation du plan Industrie du futur par Édouard Philippe

3,2 % de la richesse nationale, soit le double de la zone euro. Les investissements dans les nouvelles technologies représentaient 0,55 % de la richesse nationale en 2016, 1,2 % dans la zone euro et 1,4 % aux États-Unis. Le secteur industriel a, je vous le rappelle, madame la secrétaire d'État, mais vous le savez, un effet démultiplicateur exceptionnel en termes d'emplois et de créations de valeurs. Il y a donc urgence et intérêt à agir

Les chiffres du déclin industriel de notre pays sont connus, indiscutables et, surtout, alarmants : l'industrie française a perdu près de 1,5 million d'emplois en Alors que, en 1989, elle représentait encore 20 % de l'activité en France, elle est tombée à 12 %. Des centaines d'entreprises industrielles ont disparu, et nous avons tous été consternés par le rachat de nombreux fleurons français tels que Pechiney, Alstom, Alcatel ... Bien évidemment, nous ne sommes pas le seul pays dans ce cas-là et de nombreux facteurs entrent en jeu, comme le développement de la mondialisation et de la concurrence internationale, sans oublier l'effondrement de notre compétitivité. Ce qui est le plus inquiétant, c'est l'affaiblissement durable de notre tissu productif et notre incapacité à trouver notre place sur le marché européen et mondial. Pris en étau entre l'industrie allemande, qui fabrique des produits à haute valeur ajoutée, et les produits de gamme inférieure offerts à bas coûts par les pays d'Europe du Sud et par la Chine, nous n'arrivons pas à trouver notre place et à relever la tête. Nous avons cru aux chimères de ceux qui nous promettaient une économie désindustrialisée. Nous pensions que nous garderions, outre les emplois administratifs, que la production et la fabrication seraient externalisées dans les pays en voie de développement, comme la Chine, l'Inde ... Quelle erreur monumentale ! Quel manque de clairvoyance ! Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en mesure de nous racheter, et pas le contraire ! Alors, comment faire pour protéger, dès à présent, nos grands groupes industriels de certains prédateurs et, surtout, pour changer notre vision des choses afin de comprendre qu'il n'y a pas de grand pays sans grandes industries ? Ma question sera simple, madame la secrétaire d'État : quand la France va-t-elle enfin mettre en place une politique industrielle digne de ce nom

l'Allemagne compte autant d'entreprises de taille intermédiaire, c'est parce que celles-ci bénéficient d'un régime tout à fait particulier, totalement défiscalisé, celui des fondations.

Et nous, si nous laissions faire le marché et nous désengagions capitalistiquement de nos entreprises, nous ferions la plus grande des erreurs Faisons en sorte, justement, d'équilibrer nos rapports entre l'Europe, la Chine et l'Amérique et, surtout, faisons en sorte que la France, dans ce concert européen, joue un rôle de premier plan ! Madame la secrétaire d'État, nous avons des dossiers très importants